je vous remercie qu'il démissionnait de son mandat de sénateur de la Meurthe-et-Moselle à compter du samedi 31 décembre 2022 à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il a été remplacé par Mme Véronique Del Fabro, dont le mandat de sénatrice a commencé le dimanche 1 janvier 2023, à zéro heure. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues, la conférence des présidents a inscrit le prochain débat d'actualité à l'ordre du jour du mercredi 11 janvier à seize heures trente. Après concertation avec les groupes politiques, ce débat porterait, sur proposition du président du Sénat, sur le thème suivant La crise du système de santé », sous forme de discussion générale d'une heure. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. ainsi décidé. Sur proposition du président du Sénat et en accord avec le Gouvernement et les groupes politiques, nous pourrions fixer les explications de vote et le scrutin public solennel sur solennel sur le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes au mardi 24 janvier à

de la proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses le mercredi 1 février au soir. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Par courrier en date du 17 décembre dernier, M. Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du jeudi 2 février de la proposition de loi visant à renforcer l'action des collectivités territoriales en matière de politique du logement et de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la Première Guerre mondiale. Acte est donné de cette demande. Pour l'examen de ces deux textes, les commissions se réuniraient le mercredi 25 janvier au matin et nous pourrions fixer le délai limite de dépôt des amendements de séance au lundi 30 janvier à douze heures.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'année 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. La première victime de ce climat caniculaire, la plus discrète, mais la plus durablement touchée, c'est l'eau. C'est un lieu commun de dire que l'eau nous est vitale, non seulement au sens biologique, mais aussi au sens économique. C'est une évidence de constater que le réchauffement climatique tend à la raréfier et que notre utilisation tend à la souiller.

Dans ce contexte, les perspectives économiques et écologiques de la gestion de l'eau retiennent naturellement l'attention. En introduction à ce débat, il nous revient de rappeler les lignes de force et les principaux enjeux

et ce de manière croissante, à des coûts élevés d'entretien, de rénovation, voire d'investissement dans les réseaux de distribution. D'un côté, elles ne peuvent pas y faire face seules et leurs moyens doivent être renforcés. D'un autre côté, leur liberté se doit d'être défendue. À cet égard, le Sénat s'est prononcé, à la quasi-unanimité, sur la nécessité de préserver la souplesse d'un transfert facultatif de la compétence eau et assainissement de la commune vers les intercommunalités, ce pour une raison très simple : l'eau répond à une logique de bassin versant et non de périmètre intercommunal. Il est également une autre évidence : ce transfert, rendu obligatoire d'ici à 2026, a déjà engendré une augmentation significative du prix de l'eau pour l'usager.

sur les moyens de cette gestion locale ne saurait faire l'économie d'une réflexion précise quant aux moyens des agences de l'eau. Celles-ci constituent les principaux relais des politiques de l'eau et des programmes pluriannuels d'intervention. Leurs ressources, d'environ 2 milliards d'euros, proviennent pour 80 % des redevances des usagers. Le périmètre de leurs interventions s'élargit toutefois continuellement, y compris au-delà de la fourniture d'eau potable et de l'assainissement, jusqu'à divers investissements ayant trait au petit cycle comme au grand cycle de l'eau. Lors du débat organisé sur leur financement, ici même, au Sénat, au mois de janvier dernier, le Gouvernement a pris l'engagement de présenter les grands axes de leur renforcement, après qu'elles eurent subi l'abaissement de leur plafond de recettes en 2018 et la ponction de leur budget au profit de l'Office français de la biodiversité. Cet élargissement des actions des agences de l'eau, allié à l'écrêtement de leurs moyens, fait craindre que, contrairement au principe fondateur en vertu duquel « l'eau paie l'eau », l'eau ne paie désormais l'État. Une deuxième ligne de force de la gestion économique locale se dégage donc à son tour : les missions et les moyens des agences de l'eau nécessitent un réajustement précis destiné à sécuriser économiquement cette filière. telle sécurité économique doit par ailleurs aller de pair avec une sécurité écologique. En second lieu, l'eau doit faire l'objet d'une gestion et d'une consommation plus vertueuses. Parce qu'elle n'est pas une ressource infinie, elle doit être utilisée en conscience. Il faut le rappeler clairement : l'eau est d'abord un flux, représentant un volume de 510 milliards de mètres cubes de précipitations annuelles, inégalement réparties sur le territoire et minoritairement captées par nos cours d'eau et nos nappes phréatiques ; 35 milliards de mètres cubes y sont prélevés et 5 milliards de mètres cubes sont consommés. L'eau est ensuite un stock, naturellement contenu à hauteur de 2 000 milliards de mètres cubes et artificiellement retenu pour environ 12 milliards de mètres cubes. Pourtant, à l'heure actuelle, tous ces chiffres sont devenus faux : le réchauffement climatique nous impose de fonder nos réflexions sur des volumes diminués, sur des débits annuels amoindris et, par conséquent, sur la perspective d'une consommation rationalisée. C'est pourquoi il paraît désormais indispensable d'appliquer à cette ressource une lecture économique, permettant une action raisonnée, d'une part, sur la demande, d'autre part, Quant à la demande, d'abord, les objectifs de réduction de la consommation de l'eau, définis lors des assises de l'eau de 2019, doivent faire l'objet de pédagogie ainsi que de mécanismes incitatifs qui font actuellement L'agriculture, qui représente les deux tiers de la consommation, doit modifier en profondeur ses pratiques et se résoudre à un effort de sobriété, notamment en suivant des cycles d'utilisation plus vertueux grâce à l'optimisation technique de l'arrosage et à la récupération de l'évaporation. Quant à l'offre, ensuite, la création de moyens collectifs de retenue et de stockage d'eau nécessite d'appliquer une régulation, voire une certaine discipline, au stockage individuel. Dans le même sens, le développement de l'assainissement doit permettre d'accroître les volumes d'eau susceptibles de réutilisation après traitement, voire de recharge artificielle des nappes phréatiques. Dans tous les cas, je tiens à insister sur la nécessité d'une concertation et d'une application locale de la politique de l'eau. Seule l'association des collectivités et des communes est à même de garantir l'efficacité et l'effectivité des dispositifs de gestion de l'eau. Force est de souligner, à cet égard, l'impérieuse nécessité de poursuivre la rédaction de projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), instruments d'une sobriété localement concertée. Il y a là une condition indispensable pour que tous nos concitoyens prennent conscience de leur solidarité naturelle, laquelle doit valoir entre territoires comme entre usagers. Il s'agit également d'un critère d'équité dans la fixation du coût de l'eau, qui doit rester supportable pour tous.

Pour faire face à la raréfaction de l'eau et en concilier l'ensemble des usages, une véritable stratégie de sobriété est donc indispensable. C'est l'option la moins coûteuse et la plus efficace pour faire face aux épisodes de sécheresse. Parallèlement, il conviendra de déployer un véritable panel de solutions variées pour mobiliser la ressource. L'eau est en effet la ressource la plus précieuse du XXI siècle. La parole

dialoguer, écouter, débattre, agir : sur le sujet de l'eau plus encore peut-être que sur tout autre sujet, il nous faut faire tout cela en même temps, alors même que l'urgence climatique bouleverse notre gestion quotidienne de l'eau.

Dans un pays comme la France, l'eau est majoritairement tenue pour acquise, courante et peu chère. Toutefois, si nous voulons la préserver, nous devons lui redonner sa véritable valeur et apporter le plus grand soin à la gestion de cette ressource stratégique. Le changement climatique entraîne des bouleversements profonds du cycle de l'eau. La sécheresse que nous avons connue en 2022 a été intense et prolongée. Elle a eu un retentissement sans précédent auprès de l'opinion publique. De très nombreux Français ont ressenti ses effets dans leur quotidien, au gré des restrictions et des interdictions. Cet épisode a fait prendre conscience à nos concitoyens à quel point l'eau était une ressource précieuse et un patrimoine commun de la Nation à préserver. Il a aussi révélé des éléments à améliorer dans notre gestion de crise. Tel est l'objet de la mission d'inspection qui a été diligentée et qui rendra ses recommandations au premier semestre de 2023.

nous avons une politique de l'eau structurée, organisée et fortement outillée. La France a placé les collectivités au centre de la politique de l'eau. L'organisation par bassin fait figure d'exemple sur la scène internationale et nous pouvons, collectivement, en être fiers. Nous disposons d'outils et nous sommes en mesure de trouver des solutions face aux défis qui se présentent à nous. Je vois cette prise de conscience de l'opinion publique comme une occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs- particuliers, industrie, agriculture, tourisme, secteur public -dans une même dynamique, sans opposition, sans accusation. Si, aujourd'hui, nous reposons les termes d'un débat sur la ressource en eau, c'est parce que sa raréfaction rend la question du partage entre ses différents usages de plus en plus cruciale. Nous devrons être capables d'arbitrer la question du partage de cette ressource, dans la concertation et dans un esprit de responsabilité collective. Il nous faut aussi construire un cadre propice au déploiement de solutions dans les territoires. nous donner les moyens d'investir pour économiser l'eau, l'utiliser efficacement et selon une logique circulaire, préserver sa qualité et minimiser l'impact environnemental de cette utilisation. Je sais que le Sénat est particulièrement attentif au sujet de la gestion de l'eau. Les territoires sont en première ligne face aux enjeux et défis afférents. Je veux avoir un mot pour pour les collectivités, pour les services de l'État et pour les acteurs économiques qui ont été les plus confrontés à la gestion de crise, car je sais que cette année a été particulièrement éprouvante.

Vous vous demandez de quels moyens disposeront les collectivités pour agir dans la préservation du grand cycle de l'eau. Vous vous posez la question de la mise en cohérence des échelons de gouvernance. Vous promouvez un dialogue renforcé entre les instances de définition des politiques publiques territoriales. Vous vous interrogez sur la possibilité de lever des freins à l'innovation, dont certains sont réglementaires, comme sur le sujet de la réutilisation des eaux usées. Ces questions font pleinement écho aux enjeux identifiés lors du lancement du chantier sur la gestion de l'eau qui s'inscrit dans la planification écologique promue par la Première ministre. Christophe Béchu, Agnès Firmin Le Bodo et moi-même avons inauguré ce chantier, le 29 septembre dernier, avec l'objectif de coconstruire un plan d'action mobilisant l'ensemble des parties prenantes, de bâtir du consensus et de repolitiser le sujet de l'eau.

Nous avons ainsi mobilisé le Comité national de l'eau (CNE) pour organiser une large concertation des acteurs. Cette concertation, nous avons souhaité qu'elle soit également déployée dans les territoires, dans les comités de bassin, car notre volonté est bien d'affirmer le principe d'une politique de l'eau décentralisée et concertée avec l'ensemble des usagers. La phase de concertation vient tout juste de s'achever. Le Comité national de l'eau et les présidents des comités de bassin m'ont présenté leurs contributions jeudi Je tiens à souligner la richesse des réflexions, l'important travail accompli pour construire du consensus et les propositions très concrètes qui ont été formulées. Ce plan d'action ne sera pas le plan d'action de l'État

de qualité ; restaurer un grand cycle de l'eau fonctionnel pour préserver les écosystèmes. Ce plan traduit une conviction commune : la ressource en eau en France est précieuse, précieuse pour nos écosystèmes, précieuse pour notre santé, précieuse pour notre économie. Nous devons repolitiser les enjeux territoriaux de l'eau, en particulier les questions de partage de la ressource. Nous devons nous réunir autour d'une ambition forte pour favoriser des solutions d'adaptation dans nos territoires. Je serai ravie de revenir au Sénat vous présenter l'ambition et le contenu de ce plan. En attendant, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous allons

Concernant la rareté de l'eau, la situation devient tendue. Dans nos territoires du Sud, des communes sont régulièrement ravitaillées en eau potable. Se posent donc plusieurs questions quant à la gestion de la ressource. Comment favoriser encore davantage le partage de l'eau dans un contexte de croissance démographique ? En trente ans, la consommation d'eau a doublé à l'échelle mondiale. Il faut donc raisonner globalement. qui est de la filière agricole, l'irrigation devrait s'accompagner de formations obligatoires et de quotas par production. Quant à la consommation d'eau potable, malgré les messages de sensibilisation, elle n'est toujours pas raisonnée- songeons, par exemple, à l'utilisation d'eau potable pour laver les voitures ou alimenter

Deux axes me semblent importants. Le premier axe est de faire de la sobriété une politique publique prioritaire. Nous informerons mieux les Français sur les bons gestes.

mentionnant les retenues collinaires. Cette solution doit être étudiée au cas par cas : il n'est pas question de la généraliser en France, mais chaque projet qui respectera les critères exigeants que nous fixons pourra être validé. Nous aurons l'occasion, pendant ce débat, de revenir plus en détail sur ce sujet. La parole

Dans un contexte d'adaptation aux effets du changement climatique, des solutions sont à rechercher pour que les activités consommatrices d'eau puissent se poursuivre. Dans le domaine agricole, la réponse passe en partie par la possibilité de continuer à irriguer, même pendant les périodes de sécheresse, lesquelles, certaines années, débutent dès le printemps. Toutefois, la ressource en eau se raréfie. raréfie. Encore fortement agricole, le département des Deux-Sèvres figure parmi les plus touchés par les effets de la sécheresse. Confrontés au premier chef aux aléas liés au changement climatique, les agriculteurs deux-sévriens ont dû et ont su s'organiser pour maintenir leur production en qualité et en quantité. Réunis au sein d'une coopérative de l'eau, ils se sont engagés dans la réalisation de retenues de substitution afin d'alléger la tension sur la ressource en eau, ces réserves permettant de stocker de l'eau en période hivernale. Il convient de rappeler que ce projet a été lancé voilà une dizaine d'années, après concertation, avec l'accord des hydrogéologues, de l'État, des collectivités territoriales, des associations environnementales et des agriculteurs. Parallèlement, ces mêmes agriculteurs se sont engagés à faire évoluer leurs modes de production et se sont tournés vers des cultures moins consommatrices en eau. Le département des Deux-Sèvres est aujourd'hui tristement connu pour la manifestation violente que ce projet d'investissement a suscitée le 29 octobre dernier, notamment à Sainte-Soline. Ces investissements, pourtant autorisés, font l'objet de contestations et de sabotages. Les porteurs de projet et les entreprises sont soumis à des intimidations. Les conditions dans lesquelles les entrepreneurs interviennent s'en voient dégradées.

Les seize retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole dans le bassin versant Sèvre Niortaise et Mignon, notamment à Sainte-Soline, constituent une réponse adaptée aux enjeux du territoire, dans l'objectif d'atteindre une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. Le protocole a été validé en 2018 et signé en présence d'élus de toutes sensibilités ; je ne les nommerai pas ici, mais vous en connaissez un certain nombre. Il est soutenu par l'État pour trois raisons parce que celui-ci a proposé à tous les acteurs du territoire un cadre de concertation pour parvenir collectivement à un projet équilibré entre les besoins agricoles en eau et la préservation de l'environnement deuxièmement, parce que les réserves de substitution dans ce bassin versant sont pertinentes pour améliorer la situation durant l'été, comme cela est confirmé par les études scientifiques troisièmement, parce que le projet de réserves de substitution a été conditionné à des contreparties du monde agricole- je pense à la réduction de 50 % des pesticides, aux mesures en faveur des zones humides et de la biodiversité ou encore aux évolutions vers des pratiques agroenvironnementales et des cultures moins gourmandes en eau -, ce qui permet d'accélérer la transition écologique. Le projet, qui a été légalement autorisé, apporte des garanties nécessaires en matière de prélèvement de la ressource en eau. Les études scientifiques du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de 2022 montrent un gain de débit dans les cours d'eau et de plusieurs mètres de hauteur dans les nappes pendant la saison d'étiage ; les conditions de remplissage hivernales sont strictement contrôlées. Si les niveaux des nappes souterraines sont inférieurs aux seuils fixés par arrêtés préfectoraux, le remplissage des réserves de substitution est interdit. Soyez assuré que le Gouvernement sera très attentif à la situation du territoire

de limitation des usages de l'eau. L'état de sécheresse de cet été s'est étendu à l'automne. La question de la quantité de la ressource en eau dans notre pays se pose donc plus que jamais. D'un point économique qu'écologique, la gestion de l'eau est indispensable. Je prendrai l'exemple de l'agriculture : les sécheresses que nous connaissons depuis plusieurs années ont un impact sur notre souveraineté alimentaire. Notre agriculture perd des parts de marché aux échelons européen et international. Gérer l'eau suppose que l'on puisse poursuivre l'irrigation des terres. Qu'est-il prévu concernant les évolutions des systèmes d'irrigation et de rétention d'eau de pluie- les retenues collinaires d'hiver -en agriculture ? La gestion de l'eau est également essentielle quand il s'agit de production d'énergie des moulins ou des barrages. La petite hydroélectricité et les grandes installations sont à la croisée d'enjeux économiques, écologiques, énergétiques,

Dans l'état actuel des choses, si rien n'était fait, beaucoup de PME seraient en grande difficulté. Nous devons en effet sortir de la dépendance énergétique. Une meilleure gestion de l'eau peut y participer. La petite et la grande hydroélectricité font partie des solutions. Madame la secrétaire d'État,

je partage votre analyse : le changement climatique en cours aura un impact fort sur notre agriculture. C'est pourquoi le précédent gouvernement a engagé un Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, afin d'évoquer les solutions face à ce défi. Une feuille de route a aussi été présentée par la Première ministre au mois de mars dernier. C'est bien une dynamique d'adaptation que défend le Gouvernement, avec un panel de solutions qu'il conviendra de mobiliser. Les agences de l'eau et FranceAgriMer accompagnent financièrement l'adaptation de l'agriculture. Dans le cadre de France Relance, plus de 170 millions d'euros ont été dédiés à l'investissement dans les matériels d'irrigation plus performants, par exemple le goutte-à-goutte en arboriculture, le pilotage basse pression en grandes cultures, ainsi que les projets hydrauliques collectifs.

deuxièmement, renforcer la résilience de l'agriculture dans une approche globale, en agissant sur les pratiques agricoles et l'efficience de l'irrigation, troisièmement, accéder à une vision partagée et raisonnée de l'accès aux ressources en eau. Il faut continuer à travailler à la fois sur l'adaptation et la mobilisation des ressources. Les plans d'adaptation des filières doivent se saisir pleinement de l'enjeu de changement climatique, comme l'a fait la filière viticole. Les chambres régionales d'agriculture réfléchissent à des projets territoriaux qui seront indispensables. La diffusion des solutions doit se généraliser dans toutes les exploitations.

On a longtemps cru que, en France, son accès était garanti pour tous et pour tous les usages. Toutefois, en 2022, 80 % des départements furent soumis à des obligations de restriction, dès l'hiver pour certains d'entre eux. Les sécheresses inédites et intenses annoncent un niveau jamais atteint du bouleversement climatique, qui a touché le cycle même de l'eau. Ce n'est pas un aléa météorologique, c'est une transformation qualitative- élargissement et assèchement de la couche atmosphérique, baisse et non-reconstitution des nappes phréatiques -qui impose des changements de pratiques dans tous les secteurs : vie quotidienne, nucléaire, industrie, agriculture. Si cette dernière elle peut être aussi source de solution en s'adaptant à des cultures plus économes en eau et en favorisant le stockage carbone. Face à la raréfaction de la ressource, le partage de l'eau devient un enjeu crucial, objet de conflits, parfois dramatiques comme à Sivens avec la mort de Rémi Fraisse.

nous le jugeons nécessaire -de mieux partager la connaissance et les analyses scientifiques ? Si oui, comment ? Nous proposons, pour notre part, un doublement des crédits de la recherche. Quelle modification le Gouvernement entend-il soutenir pour le partage de la ressource en eau : évolution de l'agriculture vers l'agroécologie ? Limitation de l'impact du nucléaire ? Priorisation des usages essentiels du quotidien face aux usages superflus ou de confort ? La parole est à Mme la secrétaire d'État.

des priorités. Plus d'une centaine de collectivités se sont en effet retrouvées en difficulté cette année. Nous avons confié une mission aux inspections pour faire le retour d'expérience sur la gestion de la crise, afin d'être prêts pour la saison prochaine. Cette mission formulera des propositions qui seront évoquées avec l'ensemble des parties prenantes, réunies au sein du Comité national de l'eau (CNE). Sur cette base, nous mettrons à jour les procédures. Il s'agira de réviser le guide national sécheresse et de s'assurer de la mise à jour des arrêtés-cadres et du plan Orsec aussi demandé aux préfets d'établir la liste de l'ensemble des collectivités ayant rencontré des difficultés d'approvisionnement et d'accompagner en priorité les plus fragiles pour améliorer leur résilience d'ici à l'été prochain. Cela passe notamment par le développement des interconnexions de réseaux. Le Gouvernement engagera 100 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour les agences de l'eau. Ce n'est pas

J'ai aussi demandé que les entreprises fortes consommatrices d'eau fassent l'objet d'inspections afin que des solutions en termes d'économies d'eau et d'anticipation des restrictions puissent être évoquées avec elles. Au-delà de la gestion de crise, c'est tout un ensemble de mesures de gestion structurelle de la ressource en eau qui doit nous permettre de garantir l'adéquation entre disponibilité de la ressource et besoins des différents usages. Tel est l'objet du plan que j'ai déjà évoqué.

L'été dernier, l'ensemble de notre pays a été touché par la sécheresse, des restrictions d'usages, plus ou moins sévères, ont été mises en oeuvre. Ce fut le cas dans le Finistère. Depuis 2001, la France métropolitaine a perdu 14 % de ses ressources en eau renouvelable par rapport à la période de référence précédente.

Plus généralement, il nous faut parvenir à un consensus sur l'eau en associant toutes les parties prenantes. Cela passera par un effort de démocratisation, d'éducation, mais aussi de communication ciblée et continue sur les usages et leur priorisation.

se doit d'être plus résiliente, plus fiable, et ce dans les trois domaines principaux que sont l'industrie, l'agriculture et les usages du quotidien. Pourriez-vous nous préciser la méthodologie retenue et les actions à venir en la matière ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice Havet,

Le diagnostic est sans appel : on évalue à 81 % l'effondrement des espèces d'eau douce ; trop de territoires sont en déficit ; 30 % des eaux souterraines ne sont pas dans un bon état chimique. Nous devons donc accélérer de manière coordonnée.

renforcer la gouvernance sur son partage, garantir l'accès à une eau potable de qualité et restaurer le grand cycle de l'eau. Une des clés de la réussite passera par une planification efficace, qui conduira très rapidement à la réalisation de projets. Pour coconstruire le plan d'action, j'ai mobilisé l'ensemble des parties prenantes afin de bâtir du consensus, mais aussi de repolitiser le sujet de l'eau. Les contributions du Comité national de l'eau et des comités de bassin ont été présentées jeudi dernier. Les acteurs m'ont transmis de nombreuses propositions qui touchent à la fois à la gouvernance, aux outils réglementaires et au financement. J'examine actuellement ces propositions et je tiens à saluer la qualité du travail qui m'a été remis.

je souhaite vous alerter sur une question déterminante qui a l'avantage d'allier les deux sujets préoccupants du moment : gestion de nos énergies et gestion de l'eau. Je parle ici des barrages hydroélectriques et des lourds enjeux qu'impliquent la mise en concurrence pour l'attribution de leur exploitation et le renouvellement des concessions. Depuis quinze ans, la Commission européenne fait pression sur l'État pour obtenir la mise en concurrence des barrages hydroélectriques. La France a ainsi reçu deux mises en demeure, en 2015 et en 2019. Le choix des futurs concessionnaires ne sera pas anodin : ils auront en charge la régulation des cours d'eau, mais surtout la responsabilité de 12 % de la production énergétique métropolitaine, part importante qui fait de la France le troisième pays européen en termes de puissance installée. En cette nouvelle année, plus de 150 concessions arrivent à échéance. Nombre de parties prenantes se sont déjà opposées à la décision verticale de mise en concurrence, tant elle est éloignée des enjeux territoriaux, et soutiennent, dans un même temps, le maintien du du quasi-monopole d'EDF. L'échéance se rapproche fatidiquement et soulève de nombreuses problématiques : iniquité de la mise en concurrence avec les pays membres, pertes d'emplois, hausse des prix de l'électricité, danger pour la sûreté des usagers et la sécurité d'approvisionnement, inégalités entre collectivités.

Une telle situation nuit aux investissements dans le secteur et elle est source d'incertitude pour les entreprises, les agents, la population, mais aussi les élus. C'est dans ce contexte que le Gouvernement explore plusieurs scénarios pour le renouvellement des concessions hydroélectriques. Il sera particulièrement attentif à ce que la solution retenue permette la pérennisation et le développement du parc hydraulique français, au bénéfice du système électrique français et des emplois liés à ce secteur d'activité.

Quelle que soit la solution retenue pour la gestion des concessions hydroélectriques françaises dans le cadre de la résolution de ce contentieux, le Gouvernement sera très attentif au potentiel énergétique, technique et humain des sociétés hydroélectriques et à leur ancrage territorial. Il sera en outre, dans le contexte de l'adaptation au changement climatique, tout aussi précautionneux quant aux enjeux de gestion de l'eau. Ces enjeux peuvent notamment passer par une politique de soutien à l'étiage, à l'instar de celle qui a été menée l'été dernier pendant la sécheresse historique que nous avons connue, afin de préserver le débit de certaines rivières ou de certains fleuves, et ainsi de conjuguer les différents usages possibles de l'eau à l'aval. Ce soutien à l'étiage a conduit à utiliser une fraction de l'eau des grands réservoirs hydrauliques, non pas pour faire du turbinage à des fins économiques, mais pour apporter des volumes complémentaires dans le contexte de sécheresses.

En France, nous n'avons pas attendu la directive-cadre sur l'eau, puisque, depuis leur création en 1964, le combat quotidien des agences de l'eau est d'assurer le bon état des eaux. Érigées en six établissements publics, elles ont pour mission de lutter contre les pollutions de l'eau en garantissant la protection des milieux aquatiques. Après avoir subi des baisses d'effectifs continues, allant jusqu'à la suppression de plus de 20 % de leurs emplois, leurs moyens financiers ont été rabotés depuis 2018 ... Même avant ! ... par l'instauration du plafond mordant, qui limite leurs capacités d'interventions financières auprès des collectivités territoriales, établissements

de mise aux normes des installations d'assainissement non collectif, particulièrement onéreuse pour les usagers. Madame la secrétaire d'État, comment comptez-vous donner aux agences de l'eau les moyens d'accompagner les collectivités qui ont à faire face à ces enjeux importants à l'aune du changement climatique ?

Créées par la loi de 1964, les agences de l'eau sont un outil indispensable pour nos territoires : elles sont le bras armé permettant de mettre en oeuvre une politique de l'eau qui réponde aux enjeux des territoires.

La maîtrise du plafond des redevances contribue également à la réalisation de l'engagement pris par le Gouvernement de maîtriser la fiscalité qui pèse sur les ménages. Pour autant, nous avons trouvé des marges de manoeuvre budgétaires ces dernières années

de 50 millions d'euros pour l'année 2023 dans le cadre de la loi de finances pour répondre aux enjeux liés à la sécheresse de l'été dernier. Par ailleurs, dans le cadre du plan Eau qui sera annoncé à la fin du mois de janvier, nous préparerons les prochains programmes d'intervention 2025-2030. ne doutez pas de l'ambition du Gouvernement de doter les agences de l'eau de moyens suffisants pour répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Nous sommes rassurés ...

changement climatique, le principe selon lequel « l'eau paie l'eau » reposant essentiellement sur les seuls usagers est dépassé. La solidarité nationale doit s'exprimer.

climatique et d'une ressource en eau rare et à se partager. Les événements extrêmes que nous avons connus ont exacerbé les tensions autour de l'eau entre utilisateurs agricoles et industriels, usagers et défenseurs de la biodiversité. L'arrêt de certaines productions industrielles, la production d'électricité les centrales hydroélectriques perturbée, la perte de productions agricoles, etc. : les conséquences de la sécheresse se sont succédé et les conflits d'usages sont apparus dès lors que la priorité d'un usage sur l'autre a dû être arbitrée. Vous le savez, monsieur le président, madame d'un côté, des besoins et une demande de plus en plus importante pour l'agriculture confrontée à de fortes chaleurs, pour l'industrie du fait de la volonté de réindustrialiser nos territoires, pour la population ; de l'autre, des nappes phréatiques qui peinent à se maintenir et à se reconstituer. Cette situation entraîne des conflits d'usage, menace la cohésion sociétale et nécessite que nous nous Les usages des uns ne doivent ni pénaliser les autres ni fragiliser les écosystèmes à court, moyen et long termes. Pour cela, il nous faut aujourd'hui une gestion stratégique de l'eau, une planification globale, transversale et territorialisée de la gestion de cette ressource. À l'image des difficultés que nous connaissons actuellement en matière d'approvisionnement énergétique, n'attendons pas que les territoires entrent en tension pour mettre en place les outils nécessaires. L'anticipation et la prévention doivent guider l'action publique. Madame la secrétaire d'État, quelles sont les propositions du Gouvernement pour bâtir ce dialogue si nécessaire à la préservation du bien commun qu'est notre eau ? Que proposez-vous afin de maîtriser les conflits d'usage ? Plus précisément, que proposez-vous pour organiser le partage d'usage de l'eau, et sous quel délai ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a établi le principe de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Celle-ci relève de deux grands articles de principe. dispose que l'utilisation de l'eau et sa valorisation économique, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'article précise les différents intérêts ou usages à assurer ou à concilier. Il fixe ainsi les seules priorités légales à satisfaire : la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable. Ces grands principes doivent être respectés lors de l'examen des dossiers et l'instruction des demandes d'autorisation environnementale, y compris de prélèvement et stockage d'eau, ainsi que pour la gestion anticipée, ou de crise, de la sécheresse.

Par ailleurs, le plan Eau que nous publierons à la fin du mois de janvier comportera des dispositions en lien avec celles de la maîtrise des conflits d'usage. La raréfaction de la ressource en eau rend la question du partage entre les différents usages de plus en plus cruciale, comme vous l'avez souligné, Outre les arbitrages qui doivent être menés localement, dans la concertation et dans un esprit de responsabilité collective, il nous faut aussi construire un cadre propice au déploiement de solutions dans les territoires. Je souhaite que les collectivités territoriales se saisissent mieux de ces enjeux et que le public en soit mieux informé.

En 2022, la Bretagne a subi une sécheresse record, entraînant une pénurie d'eau durant l'été. Aussi, l'État a placé la région en alerte pendant plusieurs mois. Face à la crise, il a fallu trouver des solutions et chacun a dû être raisonnable dans sa consommation d'eau. En Bretagne se pose une difficulté majeure : le sous-sol comptant très peu de nappes phréatiques, l'approvisionnement se fait essentiellement par des eaux de surface ; or les pluies insuffisantes, la canicule estivale et l'utilisation de la ressource ont fragilisé nos réserves. Cette sécheresse a fait craindre une rupture de l'alimentation en eau potable, notamment dans les Côtes-d'Armor. La ressource, pourtant bien gérée par le syndicat départemental, s'est retrouvée fragilisée.

Face à ce constat, pour assurer l'avenir et pérenniser l'approvisionnement en eau potable, des investissements des collectivités locales sont nécessaires, voire indispensables. Quels moyens l'État a-t-il l'intention de mobiliser afin d'aider les collectivités à maintenir ce service essentiel pour les habitants, les entreprises de nos territoires et, par voie de conséquence, pour l'économie du pays ? Parallèlement, la politique de gestion de l'eau doit évoluer afin de répondre à ces nouveaux enjeux. Madame la secrétaire d'État, quelle sera votre contribution dans cette réforme plus que jamais indispensable ? Quel est, selon vous, le niveau le plus pertinent pour la gestion de l'eau : le bassin versant, la région, le département, l'intercommunalité, la commune ? Et avec quels moyens ? j'ai suivi avec beaucoup d'attention les problématiques liées à la sécheresse en Bretagne en 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor m'a alertée sur le risque de rupture d'approvisionnement en eau potable.

de sécheresse a été sérieusement anticipée : le Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (Cash) a été réuni dès le mois d'avril dernier et les préfets ont très vite reçu des instructions. Le plafond de dépenses des agences de l'eau a également été rehaussé de 100 millions d'euros, dès le mois de juin. Pour autant, nous avons été collectivement confrontés à la gestion d'une crise hors norme. Parmi les difficultés rencontrées au cours de cette gestion de crise, nous avons dû faire face à des ruptures d'approvisionnement en eau potable qui ont concerné une centaine de communes rurales. Les impacts économiques ont été difficilement supportables pour certaines filières, notamment l'élevage. Les écosystèmes ont également souffert de cette situation. Nous avons observé dans les territoires des incompréhensions en matière de gradation des restrictions et des exemptions, ainsi que des difficultés de communication. devons tirer un maximum d'enseignements de cette année historique pour affronter les futurs épisodes de sécheresse, car leur fréquence et leur intensité vont forcément augmenter. C'est le sens du travail de retour d'expérience que j'ai confié aux inspections générales des différents ministères concernés. Leur rapport, qui comportera notamment des pistes d'amélioration concrète, sera remis ce trimestre. J'ai aussi demandé aux préfets des communes qui ont connu des ruptures d'engager d'engager sans délai l'accompagnement vers une meilleure résilience pour que la situation que nous avons connue l'été dernier ne se renouvelle pas cette année. Nous savons en effet que la situation pluviométrique ne nous permettra peut-être pas de passer la saison

? Ce serait, selon moi, une bonne chose, car la question doit être traitée dans le dialogue, la coresponsabilité et la compréhension mutuelle des multiples usagers de l'eau. À l'occasion de l'évaluation du PTGE de la Midouze, les agriculteurs ont déploré la longueur et la complexité du processus.

une gestion équilibrée de la ressource en eau, de maîtriser les pressions de prélèvement à un niveau compatible avec les objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau et de répondre aux enjeux du changement climatique. L'instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l'eau a donné un nouvel élan à une gestion partagée de la ressource en eau. La démarche PTGE permet, dans une dynamique de dialogue avec tous les usagers de l'eau du territoire, d'aboutir à un programme d'action qui organise le partage de l'eau disponible dans un contexte de changement climatique. Ce programme doit mobiliser un panier de solutions : sobriété, solutions en lien avec la nature, mobilisation de nouvelles ressources, voire mesures de stockage compatibles avec l'atteinte du bon état écologique et permettant de concilier les différents usages. Faisant suite à une décision du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique a été élaborée une instruction complémentaire à celle du 7 mai 2019, qui intègre les pistes d'amélioration des PTGE identifiées par le Varenne.

Elle présente aux porteurs de projet et aux acteurs de la démarche les points fondamentaux pour sa réussite, depuis la feuille de route de cadrage et l'élaboration du programme d'action jusqu'à l'accompagnement par les services de l'État. Cette instruction détaille notamment le rôle de l'État dans chacune des étapes clés

Éléments familiers de nos paysages, ils furent un temps menacés d'une destruction intégrale par le principe de la continuité écologique, issu du droit européen, qui vise à débarrasser les cours d'eau de tout obstacle. dite Climat et résilience, est venue partiellement apporter une solution en préservant certains ouvrages d'une destruction motivée par des gains environnementaux discutables, voire négatifs. Toutefois, la Commission européenne a annoncé récemment son projet de supprimer les obstacles sur 25 000 kilomètres de cours d'eau dans l'Union européenne Ces ouvrages présentent pourtant deux avantages majeurs. D'une part, ils peuvent être considérés comme une potentielle source énergétique propre, à l'heure où l'État a pour ambition une décarbonation de sa production d'énergie. d'une source énergétique d'appoint du mix français, qui présente également l'avantage d'être non intermittente, à la différence des autres productions énergétiques renouvelables. Correspondant aujourd'hui à l'équivalent d'une centrale nucléaire, le potentiel des petites centrales hydroélectriques est encore largement inexploité. D'autre part, les récents éléments climatiques extrêmes sont venus nous rappeler que les seuils, barrages et retenues d'eau pouvaient constituer des atouts pour prévenir les inondations. Il en va de même en matière de sécheresse : lors d'une récente audition au Sénat, le directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a souligné le rôle positif des retenues d'eau dans ce domaine. Les agences de l'eau consacrent aujourd'hui d'importantes sommes à la destruction des barrages. Cet argent ne serait-il pas mieux employé s'il servait à l'entretien des barrages et à leur mise en valeur énergétique, ou encore à l'entretien des canalisations d'eau

la politique de restauration de la continuité écologique concilie les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d'eau avec le déploiement de l'hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique ou encore les activités sportives en eaux vives. Il ne s'agit en aucun cas d'une politique visant la destruction d'ouvrages sur les cours d'eau. À ce jour, la politique de priorisation mise en oeuvre par le Gouvernement a permis d'identifier les cours d'eau sur lesquels il était important d'intervenir pour procéder

La solution technique retenue consiste, selon les cas, à aménager l'ouvrage- je pense à la mise en place d'une passe à poissons, d'une rivière de contournement ou encore d'un abaissement du seuil -ou à le supprimer lorsqu'aucun usage n'est possible. Depuis 2012, environ 1 400 effacements d'ouvrages ont été recensés sur ces 11 % de cours d'eau, soit moins de 6 % des ouvrages présentant un obstacle à l'écoulement à restaurer prioritairement. Cela représente 1 % de l'ensemble des ouvrages obstacles. De nombreuses études et publications scientifiques démontrent l'intérêt d'effacer certains petits ouvrages sur les cours d'eau, tant pour la survie et la reproduction des poissons migrateurs que pour l'amélioration générale des fonctionnalités de la rivière, de sa biodiversité et de sa qualité en eau. Enfin, la politique de restauration de la continuité écologique n'a pas entravé le développement de la petite hydroélectricité, qui a progressé significativement au cours des dernières années- plus de 150 000 mégawatts supplémentaires entre 2018 et 2021 -et n'est limitée que par le faible potentiel restant.

Il pleuvra toujours autant, mais les pluies diminueront de l'ordre de 16 % à 23 % en été au profit d'épisodes plus intenses lors d'autres saisons, comme l'indique également l'étude Explore 2070. Pour dire les choses simplement, nous aurons toujours autant d'eau, mais nous n'en aurons souvent pas assez quand nous en aurons besoin et nous en aurons parfois beaucoup trop, avec des risques plus importants de crues. Bref, nous aurons de l'eau si nous savons la gérer. pouvez-vous me dire pourquoi il est vertueux et écologiquement remarquable pour un particulier de stocker l'eau de pluie dans une citerne pour s'en servir quand il en a besoin et pourquoi il n'est pas vertueux de faire exactement la même chose quand il s'agit de retenues collinaires à des fins agricoles, touristiques ou industrielles ?

nous incitent à déployer une véritable stratégie à long terme pour la gestion de notre ressource en eau. Le remède est pourtant simple : nous avons de l'eau si nous savons la garder. Créer des retenues collinaires, favoriser le stockage domestique de l'eau de pluie, améliorer l'infiltration dans les nappes phréatiques, réutiliser les eaux usées- mais on peut aussi produire de la neige ou créer davantage d'espaces végétalisés -, stocker l'eau quand il y en a trop, la garder pour la réutiliser quand il y en a moins et quand on en a besoin : c'est ainsi que nous préserverons les débits de nos cours d'eau et la biodiversité à l'étiage.

des éléments. Le changement climatique modifie d'ores et déjà le cycle de l'eau. En montagne, les chutes de neige sont de moins en moins importantes, car, on le sait, les glaciers reculent. des conséquences à la fois pour l'économie des territoires de montagne et pour tous les territoires en aval qui dépendent de cette ressource en eau. Les conséquences sont très visibles sur les domaines skiables,

En zone de montagne, l'étiage se produit en hiver, et non en été. Avec l'impact du changement climatique, de nombreuses stations de ski ont besoin de stocker de l'eau pour faire de la neige de culture et sécuriser ainsi les pistes de ski. Ces investissements ont du sens, mais il faut prévoir plusieurs points de vigilance.

n'en déplaise au Président de la République, la gestion de la ressource en eau est fortement prévisible et le récent rapport d'information de la délégation sénatoriale à la prospective démontre la nécessité de repolitiser d'urgence cette question. L'hiver que nous connaissons est tout aussi inquiétant que l'été caniculaire auquel nous avons fait face et qui n'a pas épargné le bassin de la Loire que je connais bien. En l'absence de précipitations massives dans les prochains mois, des risques de pénuries sont à prévoir. Les collectivités territoriales et les agences de l'eau sont en première ligne et se sont saisies du sujet en diligentant des études hydrologie, milieux, usages, climat (HMUC), afin d'évaluer précisément la ressource du petit et du grand cycle de l'eau pour chaque territoire. L'État ne doit pas être en retrait de cette politique publique. Des solutions de nature financière peuvent être apportées pour accroître les investissements en matière d'assainissement. La commune des Ponts-de-Cé, qui m'est familière, a la chance de bénéficier d'une usine de retraitement des eaux particulièrement performante, qui, par un procédé d'ultrafiltration, permet d'assurer une eau de très grande qualité aux usagers et un taux de fuite de l'ordre de 7 %, très inférieur à la moyenne nationale qui est de 20 %. Malheureusement, mon territoire fait figure d'exception. Aussi, madame la secrétaire d'État, prévoyez-vous un plan massif de soutien financier aux acteurs de la gestion de l'eau pour mener de front ces deux objectifs de qualité et de lutte contre le gaspillage dû à la vétusté des canalisations ? Il est un autre point sur lequel Christophe Béchu est intervenu récemment : la sobriété. À ce jour, les préfectures de département comme de région disent ne pas être outillées pour informer la population. Au regard de l'ampleur de nos futurs manques, une communication nationale est-elle prévue pour répondre à nos impératifs de gestion

secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Bigot, vous m'interrogez sur l'augmentation des coûts de la gestion de l'eau et de l'assainissement, ainsi que sur l'accompagnement des élus locaux face à cette hausse. Le financement du service public de l'eau est fondé sur deux piliers : le prix de l'eau et les subventions publiques. Le prix de l'eau a en effet augmenté ces derniers mois du fait principalement de l'augmentation du prix de l'énergie et des réactifs, comme le chlore. C'est une réalité, qui pose de sérieuses difficultés, car cela nuit très fortement à la capacité d'investissement à un moment où l'on en a fortement besoin. L'État est aux côtés des collectivités. Il faut travailler sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est d'aider les collectivités à investir. Ce sera notamment l'un des axes du plan Eau que nous présenterons d'ici à la fin du mois de janvier et sur lequel nous consultons actuellement les comités de bassin et les collectivités. La Banque des territoires sera mobilisée pour accompagner les investissements nécessaires. Le deuxième axe, c'est de limiter le coût de l'accès à l'énergie. Les mesures prises par le Gouvernement permettent de limiter fortement l'augmentation du coût de l'énergie pour les gestionnaires de services d'eau et d'assainissement, donc pour les usagers finaux. Je pense en particulier au bouclier tarifaire et à l'amortisseur, ainsi qu'au filet de sécurité. La tendance d'augmentation du prix de l'eau va continuer : elle est liée à l'augmentation des prix de l'énergie et des réactifs, ainsi qu'au coût des travaux publics. Dans les territoires où l'augmentation est très forte se pose la question de l'accès des citoyens à cette ressource. Il faudra mettre en place et renforcer les aides aux usagers les plus fragiles : je pense en particulier à la tarification incitative et solidaire. Les collectivités sont compétentes pour mettre en place une tarification sociale de l'eau.

En effet, l'obligation de ce transfert en 2026 entraîne, de fait, une perte de pouvoir de décision des élus communaux. Ces derniers mois, plusieurs propositions de loi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont visé à revenir sur cette réforme des compétences du bloc communal. Trois raisons essentielles motivent cette démarche, qui tend au maintien des compétences eau et assainissement dans les compétences facultatives des communautés de communes. Premièrement, il s'agit de garantir le libre choix des élus. La commune reste compétente en matière de distribution d'eau et d'assainissement selon le code général des collectivités territoriales. Il s'agit donc de conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale et de laisser aux communes la libre décision d'un transfert ou non.

il importe de différencier et d'adapter la mise en oeuvre de cette compétence au regard de la typologie des territoires, très variable en fonction des captages et des interconnexions existantes. La gestion de l'eau et de l'assainissement est très différente d'un territoire de plaine, de montagne, de haute montagne, de vallée, de zones humides. Elle nécessite donc une différenciation, appréciée au plus près des élus. Aussi, au regard de ces trois éléments essentiels- liberté de décision, clarification, différenciation -, le maintien des compétences eau et assainissement dans les compétences facultatives des communautés de communes permettra de satisfaire les objectifs que vous avez évoqués secrétaire d'État : limiter le gaspillage, partager la ressource, sécuriser l'accès à l'eau potable, donc décentraliser la politique de l'eau. Madame la secrétaire d'État, quelles sont les raisons et les motivations qui interdisent aujourd'hui de maintenir les compétences eau et assainissement dans les compétences facultatives des intercommunalités ?

dite NOTRe, cette obligation a depuis été assouplie avec une date limite désormais fixée à 2026. Toutefois, il ne me semble pas pertinent de donner aujourd'hui un signe de retour en arrière, car cette disposition est essentielle.

mon propos, je citerai le rapport de la Cour des comptes du mois de juin 2016, qui insiste sur l'enjeu de la rationalisation à poursuivre. La sécheresse de 2022 doit nous interpeller. Il faudra des collectivités ayant les moyens d'élaborer des projets et se placer à la bonne échelle territoriale. Par ailleurs, nous avons trouvé ces dernières années des solutions permettant d'apporter des réponses à beaucoup de problèmes locaux. Les collectivités peuvent garder un prix de l'eau individualisé par secteur lors de l'entrée dans l'EPCI. Il est possible de garder des syndicats pour assurer les compétences eau et assainissement. Ces solutions ont été élaborées et débattues avec la représentation nationale- le Sénat y a d'ailleurs beaucoup contribué. suis donc persuadée que nous avons trouvé un équilibre, qu'il faut de la visibilité et de la stabilité dans les décisions. L'enjeu maintenant est surtout d'aider les collectivités à organiser ces transferts et à investir, plutôt que de laisser penser que l'on ne peut rien changer.

À l'instar d'autres départements, l'Ardèche a souffert d'une sécheresse d'une rare intensité en 2022. Celle-ci a duré de mai à novembre et a réduit drastiquement les ressources hydriques. Ce déficit de pluviométrie a affecté tous les usages de l'eau, qu'il s'agisse des réseaux d'eau potable, de l'agriculture, de l'industrie ou des loisirs. Si des mesures de restriction ont été prises pour affronter cette crise, nous savons que cette pénurie historique et son lot de records de températures n'auront demain plus rien d'exceptionnel. Les communes et leurs groupements devront donc s'adapter à la nouvelle donne et assumer des investissements importants. Les acteurs du bloc communal déplorent déjà un désengagement des agences de l'eau,

Malgré le renfort des 100 millions d'euros fléchés vers l'investissement qu'a annoncé la Première ministre au mois de novembre dernier, les moyens de nos agences ne sont plus calibrés pour affronter les conséquences du réchauffement climatique, dont les effets se manifestent déjà. De plus, ce sont ces agences qui abondent à hauteur de 80 % le budget de l'Office français de la biodiversité, ce qui représente une ponction de 15 % de leur budget. Madame la secrétaire d'État, comment comptez-vous aider les agences de l'eau à sortir de cet effet ciseau ? ? Sans augmenter les factures d'eau des particuliers, de quelles ressources supplémentaires allez-vous les doter pour leur permettre de mener en parallèle l'adaptation des infrastructures au réchauffement et la contribution à la défense de la biodiversité ? La parole

Soyez assurée que j'ai suivi avec attention la situation de l'Ardèche. Nous devons avoir des solutions efficaces pour pallier le manque d'eau et le déficit structurel des nappes. Comme je l'ai indiqué en réponse à la question de Mme la sénatrice Varaillas, malgré l'engagement du Gouvernement à maîtriser la fiscalité qui pèse sur les ménages, nous avons trouvé des marges de manoeuvre budgétaires ces dernières années- je les ai détaillées. Je tiens aussi à rappeler que les agences de l'eau représentent presque 1 500 agents dans les territoires pour accompagner les projets. Dans le contexte que représente l'adaptation au changement climatique, j'ai été attentive à ce que ces agences disposent de moyens pour répondre aux attentes des collectivités territoriales. En termes de moyens humains, la loi de finances pour 2023 maintient, comme pour 2022, le plafond d'emplois des agences de l'eau, après dix ans de baisse. Concernant le financement de la biodiversité par les agences de l'eau, le Gouvernement entend aussi votre inquiétude. Je pense qu'il ne faut pas opposer biodiversité, grand cycle de l'eau et petit cycle de l'eau. Pour autant, je regarderai avec attention les propositions issues du rapport sur le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité pour 2030. Je vous le redis, dans le cadre du plan Eau qui sera annoncé à la fin du mois de janvier, nous devrons préparer les prochains programmes d'intervention 2025-2030 : ne doutez pas de l'ambition du Gouvernement de doter les agences de l'eau de moyens suffisants pour répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Nous sommes

après le covid-19 et la pénurie de masques, après la guerre en Ukraine et les pénuries d'huile et de moutarde, après le problème de l'énergie et l'envol des prix de l'électricité, menaçant de faire disparaître des pans entiers de notre économie-

dans votre délire catastrophiste, jusqu'à faire croire que l'eau serait une ressource épuisable et non renouvelable, comme si sa non-utilisation et le refus de la stocker permettraient de mieux se prémunir des manques à venir.

climatique pouvait laisser supposer qu'enfin vous aviez compris la nécessité de l'intérêt prioritaire de l'usage de l'eau à l'agriculture. C'était toutefois sans connaître l'obstination de notre technocratie abrutissante, qui n'aura eu de cesse, durant tous ces travaux, d'en faire au final une vraie supercherie. Alors, madame la secrétaire d'État, dans quelques années, quand les Français ne pourront plus manger à leur faim à cause des décisions que vous aurez prises, ne croyez-vous pas qu'ils chercheront des responsables ?

Alors que d'autres pays, pourtant proches de nous, comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, se sont lancés dans la réutilisation des eaux usées et dans la construction de réserves de substitution, nous continuons, nous, à regarder ces milliards de mètres cubes être gaspillés Autre preuve de la mauvaise gestion de cette ressource dans notre pays, le nombre d'acteurs qui gravitent autour de la politique de l'eau ... Le 25 janvier dernier s'est tenu dans cet hémicycle un débat sur les agences de l'eau.

Pourtant, cette mesure aurait permis de mieux financer l'eau et l'assainissement, comme l'ont rappelé Anne Ventalon, Alain Cadec et Jean-Marc Boyer.

garantir l'accès à l'eau du secteur de l'alimentation en eau potable pour les productions alimentaires. En effet, on ne peut pas continuer d'imposer aux agriculteurs d'accomplir les douze travaux d'Hercule pour pouvoir réaliser une réserve de substitution. Aux écologistes radicaux qui font le choix de la violence contre la création de ces réserves, nous devons rappeler que, jusqu'à preuve du contraire, il faut de l'eau pour l'agriculture même biologique,

Cette réforme s'impose ! Nous devons fixer un nouveau cadre- attention, pas de nouvelles normes, mais bien un nouveau cadre, plus lisible, plus accessible, pour permettre un usage efficace de cette ressource. Madame la secrétaire vous nous avez donné un certain nombre d'avis, mais je souhaite désormais que l'on transforme le verbe en actions concrètes ! Nous en avons terminé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

La population a-t-elle vraiment conscience des restrictions de circulation vouées à se multiplier sur l'ensemble du territoire d'ici à 2025 ? Non, certainement pas. Un récent sondage de l'institut Harris soulignait d'ailleurs que 60 % des sondés ignoraient même ce qu'était une ZFE

la transition écologique ne peut pas davantage s'accomplir dans un contexte de rejet social. En cherchant à « starifier » à tout crin une vision anti-voiture, vous avez omis de sanctuariser le seuil d'acceptabilité, totem de justice sociale intimement mêlé à la réussite de la mesure. À vouloir ménager un seul pan de la population, vous mécontentez tout le monde. Figés dans une sorte de sectarisme bureaucratique, vous chassez même, par l'application maximaliste

autre que la fabrique en puissance à « gilets jaunes ». C'est celle que nous avons tâché d'emprunter au Sénat. L'équilibre, ce n'est ni l'eau tiède ni le ; l'équilibre, c'est le fait de transcender les égoïsmes et de respecter le réalisme. le réalisme. « L'équilibre est un effort et un courage de tous les instants. La société qui aura ce courage est la vraie société de l'avenir »,

La ministre Pompili ne nous a pas écoutés et la majorité présidentielle a refusé nos propositions. Au Sénat, nous avons toujours défendu une écologie qui récuse les mesures strictement punitives et qui accompagne le changement. Aussi, nous avons prôné une approche territorialisée, plus souple, qui fasse confiance aux élus locaux. Le calendrier trop rapide et restrictif, faisant fi des délais réels de déploiement, impose aux collectivités territoriales un ensemble détaillé de restrictions allant à l'encontre même de la philosophie originelle de l'instrument, pensé pensé d'abord comme un outil de régulation. Nous avons proposé de revoir le schéma de restriction, de mieux prendre en compte les livraisons et le déploiement des infrastructures de recharge, de décaler la date de mise en oeuvre de l'obligation et d'assouplir celle-ci au travers d'un régime de dérogation et d'une minorité de blocage.

Nous ne mettrons pas les effectifs de police municipale pour contrôler une interdiction alors que l'État qui en est à l'origine ne mobilise pas ses propres policiers nationaux pour le faire.

Ce seul soldat sauvé est un corollaire à notre sens indispensable d'une transition juste. Plus d'un an et demi plus tard, le temps presse, mais les esprits changent. Face au mouvement bruissant de contestation, vous semblez enfin écouter nos orientations. Je vous les assène de nouveau. Dès lors que la maturité technologique des véhicules n'est pas au rendez-vous, la ZFE exclut. Dès lors que la France est encore loin de pouvoir offrir un prix de marché abordable pour les voitures propres, la ZFE exclut.

la ZFE exclut. Dès lors que les autorités organisatrices de la mobilité, étranglées par la hausse de l'énergie et sans effort partagé supplémentaire, se voient dans l'obligation d'augmenter les tarifs des billets, la ZFE exclut.

Entre les chantres de l'anti-bagnole et la suppression unilatérale de la mesure, le Sénat a fait le choix de ZFE faites avec les territoires et non contre eux. Monsieur le ministre, je vous engage donc au nom du groupe Les Républicains à poursuivre dans cette voie, en arrêtant d'imposer et en vous inspirant d'une méthode respectueuse des Français, résumée dans cette

cet outil européen, nous avons adopté, dans le cadre de la loi Climat et résilience, un calendrier progressif,

D'ici à 2025, vous l'avez dit, monsieur le sénateur Tabarot, quarante-trois agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place une ZFE et le fameux décret ayant paru pendant les vacances de Noël ne fait qu'appliquer la loi Climat et résilience en précisant les conditions normales de dérogation,

Je le répète, toutes les accélérations de calendrier procèdent de décisions territoriales et ne sont en aucun cas liées à une décision que le Gouvernement aurait soutenue, accompagnée ou justifiée. En elle-même, la ZFE ne vise pas à réduire le nombre de voitures, comme je l'entends parfois,

équivalente. Il aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute. Dans le

émissions (ZFE) soulève un certain nombre de questions, notamment pour les personnes habitant dans les territoires situés autour de ces zones. Dans les territoires peu denses, notamment dans les zones de montagne, souvent mal desservies par les transports en commun, il est impossible de renoncer à la voiture pour se déplacer et les habitants de ces à se rendre au sein des ZFE, que ce soit pour travailler, pour se soigner ou pour d'autres motifs. En outre, cela a été rappelé à plusieurs reprises, nombre d'automobilistes n'ont pas les moyens de changer de véhicule, surtout dans le contexte actuel d'inflation. On garde rarement une vieille voiture polluante par plaisir.

à ses entrées et que ces parkings soient desservis par des transports en commun performants. Cette solution, déjà évoquée dans cette enceinte, permettrait en outre de traiter le problème récurrent de l'encombrement des entrées d'agglomération. Je souhaite savoir si le Gouvernement compte proposer des aides financières aux collectivités pour ce type d'aménagements et si l'activation des ZFE pourrait être conditionnée à la présence de ces parkings relais. La parole est à M. le ministre.

connectés à des transports en commun ou à d'autres types de mobilités.

Cela implique de réduire nos émissions polluantes contribuant à la formation de particules fines. Les réflexions que nous avons échangées dans cet hémicycle sur les zones à faibles émissions furent intenses, ce qui démontre la complexité et, surtout, la nécessité de trouver des solutions efficaces.

La volonté de bien faire ne se heurte-t-elle pas aux réalités techniques et entrepreneuriales françaises ? Certaines études mettent en doute la consommation en carburant des véhicules hybrides rechargeables sur longue distance, dès lors qu'ils ont épuisé leur faible autonomie électrique.

d'une forme de souveraineté, nationale ou européenne, en réservant une partie des aides à ce qui peut être produit sur notre territoire. C'est ce que je souhaite ; je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en reparler.

du nouveau réseau express métropolitain, qui perd chaque jour en crédibilité. L'État doit peser sur la SNCF pour qu'elle réagisse rapidement. Ce dernier n'a pas tenu son engagement d'assurer aux ZFE, en 2022, un système de contrôle-sanction automatisé. Il faut se reprendre vite et bien, en assurant le retour vers les collectivités concernées de l'essentiel du produit des amendes. Ainsi, Lyon attend un calendrier et des précisions pour l'affectation de ces recettes. Ne laissons pas se décrédibiliser nos ZFE en n'assurant pas le respect des règles nécessaires qu'elles instituent.

Le contrôle-sanction automatisé ne sera pas disponible avant le second semestre de l'année 2024- je l'ai dit dès le mois d'octobre

par de plus écologiques et de faire appel à d'autres formes de mobilité, actives ou collectives, notamment avec le développement de lignes de covoiturage et de transports en commun repensés, allant des zones périurbaines aux agglomérations concernées.

Crit'Air. Relever ce défi suppose une information claire, une coordination entre les différentes zones concernées ainsi qu'un éventail d'aides et de dispositifs dédiés à la réussite de cette politique.

métropole où je vis, plus de 15 000 personnes sont exposées à un niveau excessif de dioxyde d'azote. Il y a urgence et la France est à la traîne ! Or la mise en place de ces ZFE se fait plus ou moins difficilement selon les territoires.

les véhicules des personnes en situation de handicap, qui ne sont pas concernés par le dispositif, les véhicules anciens et les véhicules utilitaires qui bénéficieraient d'exonérations. Vous

la pollution atmosphérique touche tout le monde. Les conséquences néfastes sur l'environnement dépassent d'ailleurs le cadre de nos seules frontières.

ferroviaire. En raison de la flambée actuelle du prix de l'électricité, le transport ferroviaire aurait avantage à faire rouler des locomotives diesel sous caténaire plutôt que d'utiliser l'énergie électrique.

des liaisons entre Rennes et le sud-est de la France, tandis qu'un autre projet est singulièrement avancé entre Rennes et Lille

Une fois ce constat dressé, il nous faut urgemment résoudre l'équation financière. Les dispositifs existants en matière de transition vers des véhicules propres, y compris la surprime dans les zones à faibles émissions, ne peuvent constituer une aide suffisante pour les millions de ménages modestes concernés. La diminution du prix des véhicules électriques, annoncée depuis plusieurs années, ne se matérialise que lentement ; or ce important constitue une barrière difficilement franchissable pour nos concitoyens les moins aisés. Dès lors, monsieur le ministre, ma question est très simple : comment le Gouvernement compte-t-il améliorer l'accompagnement financier des ménages les plus modestes dans l'acquisition de véhicules propres ? La parole est à M. le ministre.

attention sur le manque de lisibilité et de prévisibilité globale des ZFE-m qui handicape les entreprises et les transporteurs dans leurs décisions de renouvellement de flotte. En effet, si le cadre législatif laisse aux métropoles une grande souplesse pour déterminer le calendrier de mise en oeuvre, les conditions d'accès aux zones et les mesures d'accompagnement, cette flexibilité entraîne surtout une forte différenciation d'une métropole à une autre. Aussi, quand la majorité d'entre elles, à l'instar de la métropole bordelaise, dont je suis issue, n'en sont qu'à la phase de concertation, la métropole de Grenoble interdit dès à présent la circulation des véhicules utilitaires légers et poids lourds non classés, Crit'Air 5, 4 et 3. C'est pourquoi, en sus d'approfondir le processus d'harmonisation des mesures à l'échelon national, il est primordial que vous répondiez plus concrètement aux difficultés structurelles que rencontrent les professionnels dans leur adaptation aux nouvelles normes imposées par ces ZFE. En effet, leur parc, composé quasi exclusivement de véhicules diesel classés au mieux Crit'Air 2, est tributaire d'une offre industrielle de véhicules classés 0 ou 1 encore très réduite, notamment sur les segments des véhicules les plus lourds et ayant besoin d'une autonomie élevée. Ajoutez à cela d'importants délais de livraison, des coûts d'acquisition élevés et des incertitudes sur la disponibilité et l'avitaillement en énergies alternatives, et vous aurez autant de raisons de trouver une voie de négociation avec les métropoles afin d'obtenir des délais de mise en oeuvre. Merci de m'éclairer sur vos orientations en la matière. pouvez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, s'il est envisageable que l'État mette en place, sur le modèle de la transition énergétique des logements, différents opérateurs pouvant accompagner les entreprises, en qualité de tiers financeurs, dans leurs décisions de renouvellement des flottes ? Cette démarche incitative permettrait un recours simplifié et plus économique au rétrofitage, par exemple, mais aussi la baisse des coûts de production des véhicules Crit'Air 0 ou 1 ainsi qu'une diminution du reste à charge des demandeurs, lequel est toujours aussi élevé malgré les subventions de l'État et des territoires. La parole est à M. le ministre.

le tiers financement, je vous avoue que je m'interroge. Dans quelques jours, ce n'est pas un secret, le Gouvernement va soutenir une proposition de loi, qu'il avait appelée de ses voeux, sur le tiers financement pour la rénovation thermique des bâtiments des collectivités locales.

Le Président de la République a fait le choix, voilà quelques années, d'abandonner le projet de transfert et de maintenir l'aéroport à proximité du centre-ville. Les Nantais vont donc en subir directement les conséquences en matière de qualité de l'air dans les prochaines années. Monsieur le ministre,

réplique. Monsieur le ministre, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il allait falloir faire preuve de pédagogie pour expliquer cette réforme.

la ZFE mobilité va contraindre un grand nombre de nos concitoyens à moins utiliser leur voiture thermique, trop ancienne. S'il s'agit d'une bonne chose non seulement pour la décarbonation de notre mode de vie, mais surtout pour l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui est tout de même le but premier de ce dispositif, c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont aucun autre moyen personnel de se déplacer. C'est le cas notamment des personnes habitant dans les villes, ou en périphérie de villes, où les transports en commun et les mobilités dites douces sont à la peine actuellement.

Les services ne fonctionnent pas à plein et n'ont pas retrouvé partout le niveau d'avant-covid. Or il est légitime que tous les citoyens puissent trouver des solutions pour leurs déplacements quotidiens. Monsieur des consultations citoyennes à même d'accompagner sereinement cette transition ? Si les transports publics relèvent de la compétence des collectivités, nous savons très bien que certaines d'entre elles n'offrent pas encore toutes les alternatives utiles, faute d'investissement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire concrètement comment l'État compte aider les collectivités à court, moyen et long terme pour développer alternatives au « tout-voiture » ? Je veux parler de véritables pistes cyclables et de cheminements de piétons dignes de ce nom. Enfin, si nous voulons que le calendrier soit respecté et que l'acceptabilité sociale soit assurée,

Il faut être juste, tout n'est pas seulement de la faute des collectivités locales ou de l'offre. Le vrai sujet, c'est que nous n'avons pas retrouvé le niveau de fréquentation

les petits revenus urbains et ruraux qui se trouvent pénalisés. Où sont les bornes ? Comment les financer ? de l'aménagement des parkings extérieurs et souterrains de copropriété ? Combien de bornes de recharge allez-vous faire installer en milieu urbain et rural pour assurer la mise en conformité sans taxer les communes ? Que vont devenir les stations-service ? Va-t-on envisager, comme en Chine, des stations de recharge de batteries ?

nécessité d'anticiper les aides financières à déployer, de renforcer les mesures d'accompagnement, d'agir de manière progressive et non à marche forcée. Autant de conditions pour éviter que les ZFE, qui sont des outils pour combattre la pollution atmosphérique, ne se transforment en « en « zones à forte exclusion ». Actuellement, il demeure un reste à charge trop élevé pour un grand nombre de ménages, notamment les plus modestes, les jeunes actifs et ceux qui sont éloignés des transports en commun. Il en est de même pour les entreprises, en particulier les commerçants et les artisans, déjà fortement fragilisés par la conjoncture. attention à la césure qui pourrait s'accentuer entre les milieux urbain, périurbain et rural. En voulant laver plus vert que vert, certains territoires se dirigent malheureusement tout droit vers une ZFE restrictive et punitive. Nous avons de nombreux débats au sein de l'Eurométropole

comptez-vous faire évoluer le système des vignettes pour le rendre plus juste ?

homogène et transitoire pour les véhicules des professionnels ne disposant d'aucune solution alternative crédible.

suscite la vive inquiétude des chefs d'entreprise et artisans, qui voient se dresser devant eux un mur écologique et économique. Le durcissement des règles, entériné par le comité ministériel sur les ZFE du 25 octobre dernier, a été particulièrement mal vécu. De nouvelles restrictions d'accès aux soixante-dix-sept communes situées à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86 doivent également s'appliquer à partir du 1 juillet 2023. Elles risquent de provoquer un naufrage économique pour les 100 000 entreprises franciliennes des secteurs du bâtiment, des travaux publics et du transport routier Comment desservir les chantiers en cours, assurer les livraisons ou répondre à des marchés avec des véhicules ne correspondant plus aux critères exigés ? Vous ne pouvez ignorer, monsieur le ministre, l'absence d'offre constructeurs adaptée aux professionnels leur permettant de renouveler leur parc de véhicules utilitaires légers et de poids lourds, dans les délais impartis et à des coûts qui ne fragilisent pas leur activité. Vous ne pouvez ignorer non plus la durée d'amortissement relativement longue des véhicules destinés aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Dans ces conditions, et sans mettre en doute l'urgence à agir en faveur des populations vivant dans ces zones denses les plus polluées, il me semble nécessaire de faire preuve d'un minimum de réalisme.

Le calendrier de mise en place des ZFE sera-t-il adapté ? Des dérogations de circulation seront-elles accordées ou prolongées ? Enfin, la question des infrastructures de recharge adaptées aux véhicules professionnels reste entière. Un immense défi se pose à nous dont il faut tenir compte. La parole est à M.

ZFE vont inexorablement créer un fossé entre ceux qui pourront répondre aux normes en changeant de véhicule et ceux qui n'en auront pas les moyens et qui se retrouveront privés de l'accès aux centres urbains.

vous a posée ma collègue Elsa Schalck : comment concilier ambition écologique et progrès social pour les classes moyennes et populaires, afin qu'elles ne soient pas les victimes perpétuelles d'une forme d'écologie punitive ? L'écologie, oui, mais l'écologie pour tous !

Ce système, appliqué de manière globale, se révèle totalement insatisfaisant et particulièrement pénalisant pour les ménages aux revenus modestes et les populations les plus précaires. Faire évoluer la vignette Crit'Air devient une nécessité au moment où nombre de garagistes expliquent que certains véhicules Crit'Air 3 ou 4, bien entretenus et en très bon état mécanique,

nous trouvons ainsi face à un système qui commence à coûter très cher aux contribuables et qui ressemble à une obsolescence programmée par l'État du parc de véhicules existants. Avant d'imposer une transition brutale, ne serait-il pas judicieux de faire évoluer les contrôles techniques vers des vérifications plus approfondies des véhicules à vignette Crit'Air 3 et 4, ce qui permettrait leur utilisation dans les ZFE ?

c'est un enjeu vital, puisque la pollution de l'air réduit d'environ 2,2 ans l'espérance de vie et qu'elle entraîne plusieurs milliers de morts par an.

2023, mais c'est là encore beaucoup trop tard ! C'est en octobre 2018 que l'État et quinze métropoles se sont engagés pour développer des zones à faibles émissions d'ici à 2020. On aurait pu faire tout

équitable de cette richesse doit pouvoir faire l'objet de discussions dans le cadre d'un Grenelle des salaires. C'est un fait : la France manque de bras. Dans nombre de secteurs, les offres d'emploi restent sans réponse et les employeurs s'arrachent les cheveux.

La première des responsabilités, c'est donc de nommer correctement les maux qui traversent le monde du travail contemporain. Ce n'est qu'une fois rigoureusement identifiés qu'ils éclaireront la conjoncture actuelle. On peut communément définir la fonction première du travail comme une manière de gagner sa vie tout en contribuant à lui donner du sens. À l'inverse, quand le travail ne permet pas de vivre dignement ou qu'il se résume à des tâches dont on n'aperçoit pas la finalité, le corps social craque.

La plupart des candidats à l'emploi sont évidemment attachés au salaire, mais ils attendent aussi de leur entreprise qu'elle soit sensible aux valeurs environnementales, au dialogue social et au respect de la vie familiale. Quand cette dernière est déstabilisée par des emplois du temps découpés, des temps de transport à rallonge et des logements à prix prohibitif, le travail devient l'objet d'une longue plainte journalière et seule sa rémunération permet de le rendre acceptable. Ne nous y trompons pas, la valeur travail n'est ni de droite ni de gauche : elle est universelle, en ce qu'elle permet d'émanciper et de définir les individus dans nos sociétés modernes. S'intéresser au salaire, c'est s'intéresser aux fruits du labeur. En ce sens, le salaire est éminemment politique. Aujourd'hui, de quoi dépend le salaire ?

depuis les années 1980, la part des salaires est grignotée par des profits toujours plus importants. Ce déséquilibre croissant est susceptible d'entraîner derrière lui tout un cortège d'inégalités. En effet, en accordant une plus grande part aux profits, on favorise les détenteurs de capitaux. Nos sociétés post-industrielles tendent à exacerber cette tendance. À cela s'ajoutent certains modes de la vie moderne, qui sont de nature à créer une nouvelle économie basée sur l'intelligence artificielle, les impressions 3D, les nanotechnologies et les biotechnologies. Pouvons-nous penser que cela a un effet positif sur la rémunération des salariés ? J'ai du mal à le croire Pour bon nombre d'économistes, la robotisation de l'économie n'aurait pas nécessairement d'effets sur l'emploi et la répartition du revenu. En dépit de tous ces bouleversements macro-économiques,

À ce titre, il est révélateur que, alors que l'exécutif chante les louanges de la loi de l'offre et de la demande pour toute décision d'inspiration libérale, comme la dérégulation des salaires des grands patrons, il trouve dans le même temps révoltant qu'elle profite, pour une fois, aux salariés les moins fortunés. J'entends déjà certains pourfendeurs de l'assistanat présumé nous expliquer que notre modèle social n'encourage pas le retour à l'emploi. Je rappellerai en réponse, à toutes fins utiles, que la pénurie de main-d'oeuvre explose même dans des pays sans droits sociaux comme les États-Unis, où le a entraîné la démission de près de 5 millions de travailleurs en trois mois. Il vous faut donc quitter les postures faussement moralisatrices sur les gens « qui déconnent »- le Président de la République -et vous attaquer au noeud du problème,

À en croire ceux qui la propagent, les salaires dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est confronté de longue date à des tensions de recrutement, ont augmenté- tenez-vous bien ! -de 16 % cette année. La réalité est tout autre : dans les faits, l'augmentation réelle n'a été que de 4 %. Les principaux pourvoyeurs de cette légende sont le patronat et la majorité gouvernementale, qui l'invoquent à tout bout de champ pour contrer les critiques émises sur la stagnation des salaires dans un contexte inflationniste. Mais cela ne peut durer indéfiniment autour de l'augmentation des salaires, c'est surtout celle de la juste répartition de la richesse entre le travail et le capital et, incidemment, de l'augmentation des plus bas d'entre eux. Le cas de l'entreprise TotalEnergies Alors que le pétrolier battait un nouveau record en dégageant un bénéfice de 17 milliards de dollars, ses raffineries étaient bloquées par des salariés grévistes demandant une revalorisation salariale. un refus complet de la part de la direction. Pourtant, dans le même temps, le conseil d'administration du groupe annonçait, à la mi-septembre, vouloir « partager avec ses actionnaires les forts résultats de la compagnie » par un « acompte sur dividende exceptionnel », soit 2,62 milliards d'euros supplémentaires reversés à ses actionnaires. Le plus inacceptable dans ce conflit réside indéniablement dans le fait que la revalorisation salariale demandée par les grévistes représentait seulement 150 millions d'euros supplémentaires chaque année

à lui seul mon propos, madame la ministre, mais il est aussi symptomatique des concessions qui sont communément admises pour le capital et que l'on refuse systématiquement aux revenus du travail. Osons le dire, la juste valorisation salariale du travail est un principe cardinal au sens qu'elle représente le principal point de friction dans nos sociétés : bien plus qu'un principe d'égalité, c'est aussi le ciment de la cohésion sociale. Il est révélateur de voir que les inégalités de revenus sont, selon une étude du ministère de la santé de 2018, parmi celles qui sont les moins acceptées et vécues Cette injustice est d'autant plus mal perçue que les travailleurs français, qu'ils soient salariés ou indépendants, font partie des plus productifs d'Europe, près de quinze points au-dessus de la moyenne européenne.

Sans dogmatisme ni tabou, nous devrions pouvoir collectivement dégager les contours du Grenelle des salaires que j'appelle de mes voeux, afin que nos concitoyens puissent percevoir la transcription tangible de nos débats et que nous ne nous cantonnions pas à des postures partisanes.

à peine neuf mois après le début de la crise la plus profonde que l'Europe et le monde aient connu depuis la Seconde Guerre mondiale. De fait, l'agression russe a replongé l'économie mondiale dans de nouvelles incertitudes.

1980, ravivant le spectre d'une inflation autoentretenue par une boucle prix-salaire. C'est dans ce contexte troublé que la question du pouvoir d'achat s'est naturellement installée au coeur du débat public, ce qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur des questions fondamentales de répartition. La rémunération du travail est-elle juste et suffisante ? Le partage de la valeur, entre le capital et le travail, est-il satisfaisant ? Faisons-nous assez pour garantir que les salaires permettent une vie décente, même à ceux qui dépendent de faibles revenus ? Voilà les questions de fond qui nous réunissent pour ce débat sur l'opportunité d'un Grenelle des salaires, dans la perspective de mieux rémunérer le travail en France. Je remercie donc les sénatrices et sénateurs du groupe

minimal universel, mais aussi parce que cinq pays seulement ont instauré un mécanisme d'indexation automatique du salaire minimal, garantissant qu'il soit aussi stable que possible en termes réels, et donc en pouvoir d'achat.

Ensuite, en plus de l'inflation, le Smic est augmenté chaque année de la moitié du gain moyen de pouvoir d'achat des employés et ouvriers, de sorte à aussi prendre en compte le mouvement des autres salaires. Enfin, la revalorisation du Smic intervient tous les ans au 1 janvier, mais également en cours d'année dès que la hausse des prix depuis la dernière revalorisation atteint 2 %, ce qui permet de limiter les périodes pendant lesquelles l'inflation rogne sur le pouvoir d'achat du Smic. Ce mécanisme, auquel s'ajoutent les dispositions du code du travail sur la négociation salariale, mais aussi, parfois, d'amicales invitations du Gouvernement à négocier sur les salaires, entraîne une diffusion progressive des revalorisations. (Dares) estime ainsi qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, période pendant laquelle le Smic a connu une hausse historique, le salaire mensuel de base a augmenté de 4,4 pour les ouvriers, de 4,6 % pour les employés, et de 2,7 % pour les cadres. Rappelons ensuite que le Gouvernement a mis en place depuis le début de la crise énergétique, à l'été 2021, une série de mesures protégeant le pouvoir d'achat. L'énergie est l'un des postes de dépenses les plus contraints, qui pèse d'abord sur les ménages les plus modestes. C'est pourquoi le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire d'une ampleur sans précédent, qui a consisté à plafonner le prix du gaz et de l'électricité et à financer une prime à la pompe.

De même, l'État a allégé de 11 milliards d'euros les dépenses en énergie des entreprises. Je tiens à rappeler ces chiffres, car ils permettent de mesurer à quel point, grâce aux lois que vous avez votées au mois d'août dernier, nos concitoyens ont été protégés comme dans nul autre pays en Europe. Rappelons enfin l'existence des comités des salaires, leur utilité et la fréquence de leurs réunions. La valeur travail est au coeur de notre projet. Toutefois, si la valorisation du travail passe aussi par une hausse des salaires, soyons clairs : ce n'est pas à l'État d'en décréter l'ampleur.

L'équilibre dans la concertation est, à n'en pas douter, la méthode qui a le plus contribué à penser, à construire et à transformer notre pacte social. de l'insertion préside ainsi le comité de suivi des salaires, qui réunit chaque semestre l'ensemble des organisations patronales et syndicales pour dresser un bilan des négociations salariales dans les 171 principales branches. Le dernier a eu lieu au mois de novembre 2022. Compte tenu de la forte inflation que nous connaissons depuis plus d'un an, il a notamment visé à vérifier la conformité au Smic des minima de chacune de ces branches. Ce Ce comité démontre que le choix de la concertation est payant. Le nombre de branches qui affichent, de manière structurelle, des minima inférieurs au Smic est passé de 112 à 57 57 entre mai et décembre 2022. En novembre dernier, seules quatre branches étaient dans une situation de non-conformité depuis plus d'un an, contre une vingtaine en moyenne auparavant.

ont été autant de pierres ajoutées à notre système social si protecteur, si envié et auquel nous sommes, à raison, si attachés. Néanmoins, ce sont là des souvenirs d'un temps où l'économie était radicalement différente de celle Cette nostalgie d'un temps où l'État et les partenaires sociaux pouvaient décréter une hausse globale de tous les salaires n'est probablement pas une boussole actuelle pour les politiques publiques. À cette époque, chaque salaire était encadré par des grilles, le chômage ne dépassait pas quelques pourcents et la croissance, comme la productivité du travail, progressait chaque année à un rythme effréné. Vous pouvez certes le regretter, mais telle n'est plus notre réalité. Alors un Grenelle des salaires, pour quoi faire, mesdames, messieurs les sénateurs ? Pour instaurer un comité de suivi des salaires à côté de celui qui existe déjà ? Je pense vous avoir montré la dynamique de notre démocratie sociale décentralisée et la force et l'efficacité des actions du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. À ce stade, le Gouvernement fait le choix de poursuivre le dialogue dans le cadre du comité de suivi, dont nous observons les effets. Nous allons

est le différentiel trop important entre salaire net et salaire brut. En effet, le salaire brut engendre un coût du travail trop élevé pour nos entreprises et un salaire net trop bas pour nos salariés, ce qui ne valorise pas assez le travail. Le second réside dans la difficulté chronique des entreprises à recruter, quel que soit leur secteur d'activité, alors que notre taux de chômage demeure l'un des plus élevés d'Europe. Plusieurs causes expliquent

il existe aussi des freins au travail, qui n'encouragent pas suffisamment le retour à l'emploi. Nous avons récemment adopté un projet de loi visant à réformer l'assurance chômage.

plus le volume de cotisations augmente et plus le volume des indemnisations diminue. Je l'ai dit d'emblée, il est nécessaire de rémunérer le travail, mais cela

Quelles sont vos hypothèses de travail ? Comment accompagner une meilleure valorisation du travail dans notre pays et rétablir la valeur travail

Entre 1996 et 2020, le salaire médian, en euros constants, a augmenté de 16 %. Les revenus du premier décile et du neuvième décile ont augmenté respectivement de 18,5 % et de 19 %. C'est là aussi un signe d'adéquation entre les différents niveaux de salaires. La politique de soutien des salaires est donc pertinente. La parole

Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la ministre, cela fait deux ans maintenant que l'inflation rogne le pouvoir d'achat des Français, notamment des ménages les plus pauvres. L'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de près de 6,7 % au mois de décembre, soit plus que dans certains pays européens, comme l'Espagne.

La situation est d'autant plus intenable pour les ménages ruraux comme pour les plus pauvres que l'énergie et l'alimentation constituent des postes de dépenses plus importants que pour la moyenne des Français. Ces ménages subissent de plein fouet l'explosion des prix de l'alimentation,

dans la formation des salaires, afin de sortir la France de la déflation salariale

Tel est l'objet du comité de suivi des salaires, dont la dernière réunion, présidée par le ministre Dussopt, a eu lieu au mois de juillet dernier. À cette date, 112 branches sur les 171 suivies affichaient encore des minima inférieurs au Smic.

de réduire le nombre de branches en situation de non-conformité, passé de 143 à 57. Cela illustre bien le dynamisme de la négociation de branche, à laquelle nous sommes attachés.

Cette part de salaire semble n'être pour le Gouvernement qu'une simple marge de manoeuvre économique. Or les cotisations sociales sont essentielles au bon fonctionnement de nos caisses d'assurance collective et constituent le ciment de la solidarité intergénérationnelle dans notre pays.

Ces exonérations représentent bel et bien des baisses de salaire, qui mettent à mal notre système collectif et solidaire de protection sociale. Madame la ministre, notre système de protection sociale lié au travail mérite d'être renforcé.

dans un contexte de forte inflation, de nombreuses luttes ont lieu dans les entreprises afin d'obtenir des augmentations de salaire et de rattraper les pertes de pouvoir d'achat. Il n'est pas acceptable, dans la septième puissance économique du monde, de ne pouvoir vivre dignement de son travail. Or c'est bien ce qui se passe, madame la ministre ! Selon le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, le nombre de travailleurs pauvres en France est supérieur à un million. Rémunérés bien souvent au Smic, de nombreux salariés subissent des contrats précaires et des temps partiels imposés. Les femmes sont particulièrement touchées

j'aborderai une question qui me tient particulièrement à coeur et qui devrait être, à mon sens, une priorité nationale : la revalorisation du salaire des professeurs et des enseignants.

du métier d'enseignant, la juste reconnaissance de leur engagement et de leur place au sein de notre système éducatif.

Une négociation doit s'ouvrir avec les partenaires sociaux pour revaloriser les salaires au bénéfice des plus précaires, des emplois les plus utiles et les plus pénibles. Vous me répondrez sans doute, comme le ministre de l'économie et des finances, que cela entraînerait une augmentation de l'inflation.

2023 prolonge le bouclier tarifaire jusqu'au 30 juin 2023. La hausse des tarifs du gaz est limitée à 15 % à compter du 1janvier 2023 et celle de l'électricité l'est à compter du 1 février 2023. Ces mesures

C'est particulièrement vrai des jeunes travailleurs. C'est vrai aussi des métiers de première ligne, que nous avons tous salués pendant la pandémie, mais qui ont trop vite été oubliés depuis.

Il va de soi que le salaire est un moyen fondamental pour atteindre cet objectif, mais il ne me paraît pas être le seul. Portez-vous une conception extensive de la notion de travail ? Le travail doit-il être limité aux formes qu'on lui connaît classiquement ?

Les données publiées par l'Insee en 2022 montrent tout le chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ne citer qu'un seul chiffre, en France, en 2019, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 22 % à celui des hommes. Sans remettre en cause la bonne volonté du Gouvernement pour agir sur le sujet, et malgré la lente décrue des inégalités salariales observée depuis vingt ans, un tel constat demeure inacceptable. Outre la différence de volume de travail, les femmes étant plus souvent à temps partiel, cet écart de revenus s'explique aussi par le fait que les femmes n'occupent pas les mêmes emplois et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité. De plus, alors que le principe de l'égale rémunération des femmes et des hommes « pour un même travail » est inscrit dans le code du travail depuis 1972, des écarts de rémunération injustifiés persistent dans le secteur privé à poste équivalent et à compétences égales. Si la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré une obligation de résultat, avec la création de l'index de l'égalité professionnelle pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, force est de constater que la situation est toujours loin d'être satisfaisante. J'ajoute que ces inégalités de carrière et de salaires créent, voire amplifient d'autres inégalités, notamment au moment de la retraite, puisque les pensions de droit direct des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celles des hommes. Il me semble urgent d'envisager de nouvelles actions avec l'ensemble des acteurs économiques. Madame la ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier plus efficacement aux différences salariales entre les femmes et les hommes dans le monde du travail ? La parole

depuis plusieurs années, l'économie française est à la peine, et beaucoup de nos concitoyens éprouvent des difficultés pour s'en sortir au quotidien. Déjà, en 2018, les « gilets jaunes » alertaient l'opinion sur la paupérisation des territoires et de franges entières de la population

que le travail ne paie plus. Pourtant, ces acteurs économiques du territoire font partie de cette France qui se lève tôt et qui ne compte pas toujours ses heures, souvent dans des métiers ou des filières difficiles.

Je pense aux soignants et aux enseignants, pourtant si nécessaires, dont les métiers n'attirent plus les jeunes. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine ont conduit à des bouleversements supplémentaires qui ont des conséquences directes sur la vie quotidienne pertes de revenus, hausse du prix des énergies et des matières premières, difficultés d'approvisionnement, hausse des taux d'intérêt et restrictions sur les prêts ... Tous ces effets délétères concourent à un appauvrissement général, en particulier dans les territoires éloignés des métropoles et de leur dynamisme. On comprend d'autant mieux les attentes des Français sur les salaires et leurs inquiétudes quant à la réforme des retraites. Madame la ministre, quelles mesures sont prises par le Gouvernement pour redonner de l'espoir à tous ces actifs qui veulent pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail et, plus largement, pour réduire ces fractures françaises ? La parole est à Mme la ministre

Mme Corinne Féret. Madame la ministre, en France, les crises sanitaires et économiques se succèdent malheureusement, mettant en lumière une demande forte de reconnaissance, notamment par le salaire, de l'utilité économique et sociale de nombreux travailleurs précaires, à temps partiel et faiblement rémunérés. Alors que l'inflation galope au rythme effréné de 6 % sur un an, un sentiment de déclassement accable des millions de Français, contraints de s'en remettre à des primes, des allocations ou des chèques pour simplement survivre. Ces dernières années, le salaire des 10 % de travailleurs les mieux payés a augmenté trois fois plus vite que celui des 10 % les moins rémunérés. Légitimement, s'exprime le besoin d'un meilleur partage des richesses produites et la volonté de vivre dignement avec des salaires décents. On voit bien qu'il y a urgence à engager la revalorisation du facteur travail par l'augmentation des salaires, et ce sans avoir pour seule réponse des primes aléatoires, la défiscalisation et la désocialisation d'heures supplémentaires, les rachats de RTT ou d'autres mesures qui, au final, n'impliquent que les salariés eux-mêmes. organisée la première réunion nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur ajoutée. Le Gouvernement a clairement orienté le travail des partenaires sociaux vers les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale, d'actionnariat salarié et la prime de partage de la valeur ajoutée. salaires ? Madame la ministre, vous ne cessez de rappeler l'importance de la valeur du travail, souvent d'ailleurs pour stigmatiser ceux qui en sont privés. Nous avons parfaitement conscience qu'une augmentation générale des salaires ne se décide pas par la loi, mais relève du dialogue social, autrement dit d'échanges, d'écoute et de négociations. Ce n'est pas par nostalgie que nous en appelons à un Grenelle sur les salaires. Madame la ministre, quand engagerez-vous enfin un vrai dialogue social sur la question des salaires en France ?

Cela crée de nouvelles attentes et de nouvelles aspirations. Les assises du travail que nous avons lancées visent à accompagner ces évolutions sociétales et à réfléchir sur la place du travail et sur la manière dont il peut

C'est sur ce point que je voudrais aujourd'hui appeler votre attention, car les inégalités dans ce domaine décroissent trop lentement. En 2020, l'Insee estimait que le revenu salarial des femmes était encore inférieur en moyenne de 28 % à celui des hommes. Un peu moins d'un tiers de cet écart s'explique par des différences de durée de travail. de travail. Et la maternité continue d'interrompre ou de réduire sensiblement plus l'activité des femmes que celle des hommes. Les postes les mieux payés demeurent enfin, toujours selon l'Insee, moins accessibles aux femmes qu'aux hommes. La meilleure rémunération des femmes reste l'objectif à atteindre en priorité pour songer, ensuite, à une amélioration générale des revenus liés au travail. Il s'agit également d'une condition centrale pour de nombreuses priorités gouvernementales actuelles. lutter, par exemple, contre les violences intrafamiliales sans que les femmes, majoritairement concernées, détiennent la même indépendance économique que leur conjoint ? Comment assurer effectivement le plein emploi sans que cet objectif se réalise indistinctement pour les femmes et les hommes ? Le Président de la République a déjà déclaré grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. Les indicateurs et les constats d'inégalité se sont multipliés depuis la création de l'index de l'égalité professionnelle en 2018. Il est temps d'agir et d'exiger des résultats à la hauteur des engagements. Mieux rémunérer le travail en France ne peut pas s'accomplir sans justice sociale. L'égale rémunération des femmes et des hommes en constitue un pilier central. Quelles mesures concrètes le Gouvernement entend-il adopter afin de la favoriser ? La parole est à Mme

Beaucoup d'entre elles, notamment les TPE et PME, subissent les effets de l'inflation sur le prix des composants, des matières premières et de l'énergie. Leur situation économique ne leur permet pas de procéder à des augmentations. De nombreux économistes recommandent donc une autre voie : baisser la pression fiscale sur les entreprises et sur les ménages. Notre groupe appelle à une baisse du coût du travail, qui permettrait aux entreprises d'augmenter les salaires. Le Gouvernement ne s'est pas engagé dans cette voie, mais procède à des aides ponctuelles, comme la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Madame la ministre, pourriez-vous nous donner votre point de vue et nous préciser si vous souhaitez faire évoluer cette situation ? La parole est à Mme la ministre ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, le Gouvernement privilégie la confiance dans le dialogue social et les négociations salariales qui s'inscrivent dans un cadre garantissant garantissant la mise en oeuvre des mécanismes protecteurs de revalorisation du Smic. Il privilégie également l'attribution de la prime d'activité. Depuis le 1 octobre 2021, le Smic a été revalorisé à cinq reprises, au total de près de 10 %- 9,71 % -, soit bien plus

de blocage structurel. D'autres outils sont également à la main des entreprises pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Ainsi, la prime de partage de la valeur (PPV) a été pérennisée dans la loi du 16 août 2022 portant mesures 245 137 établissements ont versé 2,43 milliards d'euros de prime PPV entre le mois d'août et le 21 décembre 2022. En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'exonération des cotisations et contributions patronales pour les entreprises accordant une revalorisation d'au moins 10 %.

ma question portera sur le niveau de revalorisation et, plus précisément, sur les conclusions du rapport publié au mois de novembre dernier par le groupe d'experts sur le Smic, qui a alerté sur les conséquences négatives que pourrait avoir une plus forte augmentation du salaire minimum.

Enfin, une forte revalorisation du Smic contribuerait au tassement de la hiérarchie des salaires, entraînant une frustration légitime chez ceux qui se voient rattrapés par le Smic. Plus généralement, les auteurs du rapport expliquent que le problème n'est pas tant le niveau élevé du salaire minimum que le fait que les salaires progressent plus vite que la productivité. L'augmentation des coûts de production du fait de la hausse des salaires conduirait les entreprises soit à réduire l'emploi, soit à augmenter leurs prix de vente, et, partant, à perdre en compétitivité-prix, ou encore à réduire leurs marges, ce qui pénaliserait leur capacité à investir et à innover. Madame la ministre, pourriez-vous nous faire part de votre analyse à partir de ces recommandations ? en effet les avoir suivies, en appliquant la règle d'indexation classique pour la revalorisation du Smic en début d'année sans coup de pouce supplémentaire. Ce positionnement pourrait-il évoluer si l'inflation continue à augmenter en 2023 ? ailleurs, le groupe d'experts recommande de modifier la formule de revalorisation du Smic. Parmi les pistes envisagées, il suggère d'indexer automatiquement ce dernier sur la moyenne des évolutions de minima salariaux d'un panel de branches représentatives. Ce changement renforcerait le rôle de la négociation collective et responsabiliserait ainsi les partenaires sociaux dans la définition des normes salariales et des minima de branche. Qu'en pensez-vous, madame la ministre ?

Par le jeu des négociations collectives et des revalorisations des grilles salariales consécutives aux augmentations du Smic, les hausses se transmettent aux ouvriers et aux employés. En septembre 2022, la hausse de salaire des ouvriers et employés était d'environ 4,5 %, contre 2,7 % pour les cadres.

Des revalorisations interviennent également en cours d'année, dès que l'inflation dépasse 2 %. Ainsi le Smic a-t-il été revalorisé trois fois en 2022, deux hausses exceptionnelles ayant eu lieu le 1 mai et le 1 août Si ces revalorisations sont nécessaires pour le pouvoir d'achat des salariés et s'inscrivent dans une logique législative, leurs modalités ne sont pas sans conséquence, aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour les branches professionnelles. À l'occasion de la publication du dernier rapport du groupe d'experts sur le Smic, plusieurs organisations représentatives des entreprises ont évoqué, dans leur contribution au rapport, les difficultés liées au rythme accéléré des revalorisations du Smic. Les TPE, PME et les entreprises les plus fragiles, actuellement de grandes difficultés, voient leur masse salariale augmenter de manière imprévue et pérenne. En outre, la question de l'inflation percute le temps nécessaire aux entreprises et aux branches pour mener des négociations salariales viables et apaisées pour l'ensemble de la grille. Dans le contexte inflationniste actuel, l'application automatique du seuil de 2 % de l'indice mensuel des prix à la consommation pour revaloriser le Smic en cours d'année oblige les branches à engager de nouvelles négociations sur les salaires peu de temps après que la dernière négociation s'est terminée. Pour endiguer le phénomène, certains proposent de rehausser le seuil de l'indice mensuel à 3 % par exemple, afin de moins perturber le déroulement des négociations salariales et ainsi de laisser toute sa place au dialogue social. L'espacement des augmentations automatiques du Smic permettrait selon eux des négociations plus qualitatives dans les branches, lorsque la grille de salaires minima est impactée par l'augmentation du Smic. Il faut conclure ! Madame la ministre, que pensez-vous de cette proposition. Envisagez-vous, d'une manière plus générale, de réformer les modalités d'indexation du Smic, comme le recommande le groupe d'experts ? La parole

Elle intègre également la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés. Nous sommes ainsi l'un des cinq pays dont le salaire minimum est indexé sur l'inflation

les fermiers et les anglais rivalisèrent d'efforts pour faire descendre le salaire à son minimum absolu. À cet effet, on payait moins que le minimum sous forme de salaire et on compensait le déficit par l'assistance paroissiale. Madame la ministre, nous vivons de nos jours une situation analogue. Votre gouvernement imagine régulièrement de nouveaux dispositifs pour compenser les salaires trop bas. les salaires trop bas. La prime d'activité, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et, dernièrement, l'indemnité inflation font partie intégrante de cet arsenal. Par la prééminence de tels dispositifs, vous entretenez une situation dans laquelle les montants des salaires sont insuffisants pour vivre et où les travailleurs sont de plus en plus soumis à la contingence des aides. Force est de constater que nous ne parlons pas du même dialogue social. Nous vous parlons salaire ; vous nous parlez primes. primes. Je rappelle que la rémunération annuelle nette d'un salarié payé au niveau du Smic se répartit désormais en 84 % de salaire et 16 % de primes de pouvoir d'achat versées par l'État. Ces primes représentent l'équivalent d'un treizième mois, d'un et même un peu plus. Autant d'éléments de rémunération qui devraient être du salaire. Par ces dispositifs, l'argent public vient substituer des revenus à des salaires. salaires. Cette stratégie est une aubaine pour les entreprises : à court terme, leurs salariés touchent plus, pour un coût maîtrisé ; à long terme, les salaires restent bas. Mais il y a des perdants. Ce sont les travailleurs, qui, eux, perdent sur presque tous les plans. En effet, leurs revenus deviennent imprévisibles. Je rappelle qu'une aide distribuée par l'État peut s'arrêter à tout moment, alors qu'un salaire ne peut être baissé de façon unilatérale par l'employeur. Par ailleurs, leur progression salariale de carrière est ralentie. Enfin, pour la double peine, ils cotisent moins pour leur retraite, car ces revenus ne sont pas soumis à cotisations sociales. Ce constat sans appel ne se limite pas, tant s'en faut, au secteur privé. Aux côtés du salaire, diverses primes et indemnités plus ou moins individualisées occupent désormais une place importante dans la rémunération des fonctionnaires. Elles représentent un quart de leur rémunération et permettent à l'État de compléter un salaire qui n'augmente plus.

Qu'il s'agisse de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou de l'indemnité inflation, les primes de pouvoir d'achat ont en commun de considérer les travailleurs comme des êtres de besoins et de les réduire à cette condition. La question de la satisfaction de nos besoins, notamment matériels, est importante et même incontournable. Mais sommes-nous seulement des êtres voués à dépenser ce qui nous est accordé de façon contingente sur un marché de biens et services dont la maîtrise nous échappe totalement ? Le salaire ne se limite pas à cette considération. Tel qu'il s'est construit au cours du XX siècle, le salaire permet de reconnaître le travailleur, qu'il soit en emploi ou hors emploi, comme un producteur de valeur économique. Il n'est pas étonnant, en ce sens, que les revendications salariales se mêlent souvent aux revendications entourant les conditions de travail. Notre pays n'y coupe pas. Plusieurs mouvements de grève revendiquant une augmentation des salaires se sont enclenchés à l'automne et à l'hiver 2021, y compris dans des secteurs peu enclins aux grèves. Nous avons pu ainsi constater de fortes mobilisations dans plusieurs enseignes de la grande distribution. revendications d'augmentation générale des salaires de l'ordre de 5 %, les employeurs ont répondu par des propositions d'augmentation de 1 % ou 2 % et par des mesures contournant le salaire : doublement de l'indemnité inflation, versement de primes ou encore augmentation des remises en magasin. C'est factuel : les primes sont devenues des éléments importants de rémunération pour les titulaires de bas salaires. Finalement, les travailleurs qui mettent en valeur un capital dans le secteur privé se paient de plus en plus eux-mêmes en tant que contribuables. Cela n'est pas admissible. Dans ce contexte et alors que la période de négociations annuelles obligatoires commence ce mois-ci, j'appelle à ce que nous convoquions un Grenelle des salaires réunissant les organisations syndicales et patronales, afin qu'une réponse systémique et collégiale soit apportée aux travailleurs de notre pays. je vous remercie

territoire et du développement durable, ont saisi le président du Sénat d'une demande de constitution d'une commission spéciale sur cette proposition de loi. Cette demande a été affichée et notifiée au Gouvernement, ainsi qu'aux présidents des groupes politiques et des commissions permanentes. Elle sera considérée comme adoptée sauf si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, soit à l'ouverture de la séance du jeudi 12 janvier, le président du Sénat est saisi d'une opposition par le Gouvernement ou par le président d'un groupe.